Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui d'une proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. L'école concentre beaucoup de convictions, de passion et d'émotions, parce qu'elle est un enjeu de société, un enjeu pour les familles et un enjeu pour chaque enfant. Mes chers collègues, l'école est comme la loi : il ne nous faut la « toucher que d'une main tremblante Si la liberté d'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui inclut le droit des parents à choisir l'instruction de leurs enfants, cette liberté doit se conjuguer avec le droit de l'enfant à l'instruction, garanti par le préambule de la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Aussi, si la main doit trembler sur l'évolution de cette liberté, elle doit être ferme pour protéger les enfants de la République. La presse a ses marronniers, à savoir des sujets que l'on voit régulièrement ressurgir. La liberté d'enseignement est, en quelque sorte, un marronnier pour les législateurs, car elle est régulièrement mise en débat. Ici même, voilà plus d'un siècle, le 17 novembre 1903, le Sénat examinait le projet de loi Chaumié, qui avait déjà pour objet de substituer, à un régime d'autorisation préalable, un régime de déclaration. Permettez-moi de citer l'un de nos plus illustres prédécesseurs sur ces travées, Georges Clemenceau, qui s'adressait ainsi à ses collègues : « Vous avez fait la liberté de la presse, vous avez fait la liberté de réunion [ ...]. Vous aurez le courage de faire la liberté d'enseignement ». En 2016, dans le cadre du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, le gouvernement de l'époque avait proposé de substituer, au régime de déclaration, un régime d'autorisation préalable.

que le constat d'impuissance des autorités publiques, alors exprimé par notre éminent collègue le ministre Patrick Kanner, était incontestable et largement partagé. C'est cet amendement, déposé par mes soins en qualité de rapporteur, qui est examiné aujourd'hui sous la forme d'une proposition de loi. La liberté est indissociable de la responsabilité. D'abord, la responsabilité de l'État, qui doit veiller à l'exercice de cette liberté dans le cadre de la loi et qui doit veiller tout autant à protéger les enfants contre l'endoctrinement, l'amateurisme, l'insuffisance pédagogique, les phénomènes sectaires, voire de radicalisation religieuse. Ensuite, la responsabilité de tout établissement, qui qui doit répondre aux obligations d'instruction et d'acquisition du socle commun de connaissances, tel que défini par la loi. Quelle est la situation aujourd'hui ? L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire relève d'un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l'enseignement dispensé : premier degré, second degré général ou enseignement technique. Ces procédures ont été définies par trois lois datant du XIX siècle et du début du XX siècle. Détaillées dans une circulaire de juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, et de manière différente, le maire, l'autorité académique, le préfet, ainsi que le procureur de la République. Ces derniers peuvent s'opposer à l'ouverture d'un établissement hors contrat seulement pour des motifs liés aux bonnes moeurs- du XIX siècle -et à l'hygiène et, pour le seul enseignement technique, pour des considérations d'ordre public.

Le nombre d'élèves scolarisés dans le secteur privé hors contrat s'élève à 73 000, dont 57 % dans l'enseignement primaire relevant de la scolarité obligatoire. La progression du nombre d'établissements hors contrat est extrêmement significative : nous passons de 803 en 2010 à 1 300 en 2017, soit une croissance de plus de 60 %. Cette augmentation s'explique par divers motifs : un engouement pour des pédagogies alternatives, parfois le choix d'une éducation religieuse, une volonté d'accorder plus de place aux langues étrangères ou régionales, mais aussi, il faut le reconnaître, parfois une déception à l'égard de l'éducation nationale. L'actualité récente vient illustrer les difficultés et la zone grise juridique auxquelles nous sommes confrontés. Je pense notamment à l'école Al-Badr, à Toulouse, dont plusieurs membres de l'équipe étaient fichés S. Le procureur de la République, le préfet, le maire se sont trouvés totalement dépourvus face au refus d'obtempérer à la décision de fermeture, après un jugement du tribunal correctionnel. Le directeur d'établissement a ouvert un nouvel établissement, sous un autre nom, dans les mêmes locaux, avec les mêmes enseignants, et l'opposition de la rectrice contre cette nouvelle ouverture a été jugée illégale par le tribunal administratif de Toulouse. On peut aussi évoquer un rapport d'inspection, non publié, de 2016 de l'académie de Versailles faisant état « d'inquiétantes dérives » et de « faillite éducative ». Il est La vigilance s'impose sur les effets d'une éducation qui impose des croyances ou des convictions et occulte des pans entiers du savoir au profit d'une idéologie ». Ainsi, peut-on enseigner que Pétain a sauvé la France en 1940 ? Le législateur peut-il fermer les yeux sur des déviances qui contreviennent aux lois de la République et à la protection des enfants ? Que disons-nous à ce maire de la commune de Raismes, dans le Nord, qui ne cesse d'alerter les pouvoirs publics, mais que la loi laisse totalement seul dans le désert de ses responsabilités ? La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à simplifier, harmoniser les procédures et mieux encadrer le régime de déclaration. L'article 1 simplifie la législation, en fusionnant les trois régimes existants. Il renforce la capacité de contrôle exercée par les différentes autorités, y compris le maire, en allongeant les délais d'opposition et en unifiant les motifs d'opposition. en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s'opposer pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, et, aux services de l'État, en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants. Les sanctions en cas d'ouverture d'un établissement en dépit d'une opposition sont renforcées et le directeur académique peut mettre immédiatement les parents d'élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement. Par voie d'amendement, nous proposerons une simplification supplémentaire de la procédure, à travers l'instauration d'un guichet unique pour le dépôt des déclarations, ainsi qu'une harmonisation du délai pour toutes les autorités publiques. L'article 2 affirme le principe d'un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat. Toutefois, toutes les observations recueillies laissent à penser qu'un contrôle annuel disperserait les moyens alloués. Aussi sera-t-il proposé un contrôle obligatoire lors de la première année, avec confirmation de la possibilité, qui existe déjà, de contrôles inopinés. Monsieur le ministre, le sujet du contrôle est très important. Il conviendra de professionnaliser ces contrôles, afin d'aider les inspecteurs dans cette mission parfois très délicate, comme l'académie de Versailles l'a initié. Les inspecteurs doivent être particulièrement sensibilisés aux méthodes pédagogiques alternatives, mais aussi à l'apprentissage de certaines langues étrangères dans lesquelles se déroulent les enseignements. Cet article prévoit également que les services de l'éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public. l'article 3 étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d'âge, de nationalité et de capacité qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique. est établie, pour le directeur d'un établissement d'enseignement du second degré privé, d'avoir exercé pendant cinq ans, au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire de même type. Pour conclure, je veux saluer avec sincérité, quel que soit le vote final de leurs membres, tous les groupes politiques du Sénat pour avoir accepté de dialoguer sur ce texte, chacun dans le respect de ses convictions. Je remercie le groupe centriste, tout particulièrement son président, Hervé Marseille, qui a choisi d'inscrire ce texte dans une niche du groupe, prouvant ainsi sa conviction quant à la nécessité et l'urgence d'agir.

Mes chers collègues, ce texte est difficile, sensible- inflammable, ai-je même lu -parce qu'il touche au creuset de la République, l'école, et donc à nos convictions. Les commentaires, enthousiastes, fort créatifs de toutes celles et de tous ceux qui s'opposent à ce texte, le qualifiant de liberticide, funeste, soviétiforme, auront certainement contribué à enrichir notre vocabulaire dans la catégorie « excès de langage ». Qu'ils en soient ici remerciés ! En même temps, d'autres jugent ce texte timide, frileux, insuffisant. La contradiction de ces épithètes me semble prouver que ce texte n'obéit aux ordres de personne, d'aucun lobby, d'aucune idéologie, et qu'une avalanche de mails procédant d'une même indignation ne saurait asphyxier ou endormir la capacité des législateurs que nous sommes. Parce que nous sommes ici, au Sénat, la chambre de la sagesse, de la raison et de la réflexion, nous ne pourrons pas dire un jour que nous ne savions pas. Cette proposition est un texte de raison, au service de la République. Il n'est que cela ! Il appartient maintenant à chacun de nous, en conscience, de se prononcer sur sa volonté, par cette proposition de loi, de faire un pas pour la République et pour tous ses enfants. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel répond à un constat simple le régime d'ouverture des écoles privées est dépassé, incohérent et, à bien des égards, dangereux. Héritage de lois anciennes- loi « Falloux » de 1850, loi « Goblet » de 1886 et loi « Astier » ce régime se décline en trois procédures distinctes selon que l'établissement relève du premier degré, du second degré général ou du second degré technique. Ces procédures font intervenir, à chaque fois de manière différente, le maire, l'autorité académique, le préfet, ainsi que le procureur de la République. Elles sont rendues largement inopérantes par les délais extrêmement brefs accordés aux autorités compétentes- huit jours pour le maire, un mois pour les services de l'État -pour s'opposer à l'ouverture de l'établissement. Le caractère fortement restrictif des motifs pour lesquels il est possible de formuler une opposition contribue aussi à rendre ces régimes inopérants. Pour le premier et le second degrés, les autorités compétentes ne peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement que pour des motifs liés aux bonnes moeurs et à l'hygiène ; l'ordre public et la nature de l'enseignement dispensé sont pris en compte pour le seul enseignement technique. Curieusement, il est impossible de s'opposer à l'ouverture d'un établissement en s'appuyant sur des critères qui permettent d'ores et déjà de demander sa fermeture Ainsi, même s'il ressort du dossier que le directeur ne respecte pas les conditions d'exercice ou qu'il a été condamné pour crime ou délit contraire à la moralité, les autorités ne pourront s'opposer à l'ouverture. Or une fois l'école ouverte, seul le juge judiciaire peut prononcer sa fermeture en cas de méconnaissance de la procédure d'ouverture ou de manquement répété dans l'enseignement dispensé. Trop souvent, les maires et les services de l'État sont donc placés dans une situation de fait accompli. Le caractère obsolète des dispositions actuelles a été mis en lumière par la forte croissance de l'enseignement privé hors contrat. Le nombre d'établissements a crû : 800 en 2010, 1 300 en 2017. L'engouement que connaît le secteur privé hors contrat concerne essentiellement le primaire. En effet, tandis que les effectifs d'élèves dans le second degré régressent légèrement, le nombre d'élèves dans le premier degré a presque doublé sur la même période. Au total, le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements hors contrat a augmenté de 23 % depuis 2012, pour atteindre 73 000 à la rentrée de 2017. Contrairement à ce que certains affirment, l'objet de ce texte n'est pas de freiner ou de combattre la croissance de ce secteur. Celle-ci découle d'un phénomène de société, aux causes multiples. Je citerai plus particulièrement la défiance vis-à-vis de l'école publique, voire de l'enseignement privé sous contrat, et la préférence pour des pédagogies alternatives ou plus bienveillantes. En revanche, la multiplication des ouvertures d'établissements- 130 en 2017 -donne au problème du régime juridique une acuité nouvelle, ce que confirment certains exemples récents, comme à Toulouse. Pour autant, s'il est nécessaire d'agir, je conviens qu'il faut le faire avec prudence. Lorsqu'il détermine les règles relatives à l'ouverture des établissements d'enseignement privé, le législateur doit concilier deux principes juridiques d'égale valeur la liberté de l'enseignement- principe fondamental reconnu par les lois de la République -et le droit à l'éducation des enfants. Au-delà des seules considérations juridiques, il importe de trouver un équilibre entre l'exigence nécessaire à la protection des enfants et la facilité d'ouverture d'une école. Placer la marche trop haut risquerait de reporter une partie des projets d'école vers l'instruction dans la famille et, dans certains cas, vers des écoles clandestines. C'est parce qu'il y voyait une atteinte disproportionnée à la liberté de l'enseignement que le Sénat s'était opposé, en 2016, au projet du gouvernement de l'époque d'instituer un régime d'autorisation préalable pour l'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés. privés. En réponse à ce projet, notre collègue Françoise Gatel, alors rapporteur du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, avait déposé un amendement, dont la proposition de loi examinée aujourd'hui reprend les termes. Il s'agissait de démontrer qu'il était possible de conserver un régime déclaratif tout en l'actualisant et le sécurisant., le Conseil constitutionnel censura l'article adopté dans la rédaction gouvernementale, du fait de l'imprécision de l'habilitation à légiférer par ordonnance. Le problème reste donc entier : un régime juridique dépassé, incohérent et inopérant. C'est tout à l'honneur de notre collègue de ne pas s'être contentée d'une « victoire » juridique, mais d'avoir cherché à résoudre le problème à l'origine de ce débat. Françoise Gatel vous a présenté les grandes lignes de sa proposition de loi. Sans anticiper l'examen des articles, je souhaite évoquer les axes principaux des évolutions proposées : l'harmonisation et la simplification, d'une part, le renforcement de l'effectivité du contrôle, l'harmonisation et la simplification. Il ne faut pas moins de treize pages de circulaire pour décrire le droit en vigueur, tant les conditions diffèrent pour chaque type d'établissement. Cela est source de complexité et de confusion pour les citoyens, comme pour les maires et les services de l'État. C'est pourquoi l'article 1 de la proposition de loi tend à unifier les trois régimes d'ouverture et à mieux les encadrer, par l'allongement des délais d'examen et en permettant au maire et à l'État de s'opposer sur le fondement de l'ordre public ou du non-respect des conditions d'exercice du demandeur et du directeur. J'ai souhaité pousser cette simplification plus loin encore, en proposant la fusion des deux déclarations existantes et la création d'un guichet unique auprès des services de l'éducation nationale. Il s'agit également de distinguer clairement la personne qui ouvre l'établissement- le président de l'association qui en sera le support, par exemple -de la personne qui le dirigera. Les textes en vigueur entretiennent une confusion préjudiciable à la clarté du droit. La même exigence de simplification et d'harmonisation a présidé aux modifications que nous proposons à l'article 3. Dans le droit en vigueur, les conditions pour diriger un établissement privé et y enseigner varient fortement selon la nature de l'établissement. Elles sont particulièrement réduites pour le premier degré et, pour les enseignants du second degré général, il n'existe absolument aucune condition d'âge, de nationalité et de diplôme. À l'inverse, elles sont beaucoup plus contraignantes pour les établissements techniques. Ces disparités, si elles ont une justification historique, n'apparaissent plus pertinentes aujourd'hui, d'autant que c'est à l'école primaire et au collège que la conscience des enfants est la plus fragile et qu'il convient de les protéger. C'est pourquoi nous vous proposons, à l'article 3, une unification ambitieuse des conditions d'exercice des directeurs et des enseignants. Il s'agit d'une demande forte des principaux acteurs du secteur, qui sont confrontés à la diversité des statuts et des exigences, en particulier dans les établissements regroupant plusieurs niveaux d'enseignement. Second axe principal de notre réflexion

Or ce contrôle est encore insuffisant aujourd'hui. Les académies les plus concernées reconnaissent que de nombreux établissements hors contrat n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle. Trop peu d'établissements nouvellement créés sont contrôlés au cours de leur première année d'exercice : moins de la moitié sur Nous sommes bien en deçà des objectifs fixés par la circulaire du 17 juillet 2015, à savoir un contrôle lors de la première année et de la cinquième année d'exercice. nous ne vous proposons pas de prévoir que la loi prescrive davantage qu'un contrôle obligatoire lors de la première année d'exercice, ce qui semble être une exigence minimale. Le droit ne saurait saisir entièrement la réalité de l'action publique et du contrôle. À être excessivement prescriptifs, nous risquons de supprimer les marges de manoeuvre des rectorats et,, de limiter l'efficacité des contrôles. En la matière, rien ne remplace la volonté du ministre, volonté sur laquelle nous comptons. Enfin, lorsque des manquements sont constatés, les procédures sont insuffisamment claires et opérationnelles, du fait, notamment, d'ambiguïtés de rédaction. Mes chers collègues, je vous invite à adopter les amendements présentés par Françoise Gatel, qui reprennent ceux que j'avais présentés en commission. Ils sont l'aboutissement d'un travail de compromis visant à instituer un régime le plus simple et le plus efficace possible, conforme à l'intérêt général.

nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi de Mme la sénatrice Françoise Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. Je tiens tout d'abord à saluer cette initiative sénatoriale, qui me semble importante, car elle est à la croisée de droits et libertés qui sont parmi les plus précieux : la liberté d'enseignement, mais aussi la nécessité de protéger chaque enfant de France en lui permettant de s'épanouir dans le cadre des principes de la République. Le Gouvernement partage pleinement la nécessité de légiférer sur la question de l'ouverture des établissements hors contrat.

complexe pour les quatre administrations qui sont chargées de suivre l'ouverture des écoles avec des moyens d'action très différents entre les services municipaux, les services académiques, les services de la préfecture et ceux du procureur de la République complexe aussi pour ceux qui veulent ouvrir une école. Il est donc très important de clarifier, de simplifier et de préciser, pour sortir d'un régime obsolète, obsolète, car le régime d'ouverture des établissements privés d'enseignement scolaire qui figure au code de l'éducation résulte de la juxtaposition de dispositions de trois lois, lois, anciennes et respectables, mais qui, pour certains de leurs aspects, sont aujourd'hui dépassées : la loi Falloux du 15 mars 1850 sur l'enseignement secondaire ; la loi Goblet du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire ; la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique. Ces dispositions, codifiées en 2000, ont en commun de prévoir un régime déclaratif pour l'ouverture d'un établissement. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, très attachés aux grandes lois de la Troisième République qui portent sur l'école et sur la liberté, car elles sont nées en même temps que les grandes lois qui fondent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République- la liberté d'association et la liberté de la presse, par exemple -et notre contrat social républicain.

ce qui suppose de leur apporter les nécessaires évolutions pour qu'elles continuent à être le cadre de la vie collective et demeurent pertinentes. Aujourd'hui, le cadre juridique répond difficilement à la hausse exponentielle des ouvertures d'établissements hors contrat le rappelle à mon tour, on comptabilisait environ 800 établissements hors contrat ; aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 1 300. Cette hausse des effectifs concerne essentiellement le premier degré. Bien sûr, nous pouvons nous féliciter, sous un certain angle, de la croissance de ces nouvelles initiatives, car elles peuvent correspondre à une dynamique pédagogique qui nous montre à quel point l'éducation est un sujet au coeur de la vie des Français, que la créativité pédagogique est très dynamique en France et que la liberté d'enseignement est une réalité. une réalité. Ces principes sont évidemment respectables. Ces chiffres traduisent aussi la nécessité de moderniser et de simplifier le cadre juridique dans lequel cette liberté d'enseignement s'exerce. Du point de vue de la complexité, pour le premier degré, le second degré et l'enseignement technique, il existe trois procédures différentes avec, à chaque fois, des moyens d'action différents pour le maire, l'autorité académique, le préfet et le procureur de la République. Pour le premier degré et l'enseignement technique, une double déclaration est nécessaire auprès du maire et des services de l'État, alors que cette double déclaration n'est pas nécessaire pour l'enseignement secondaire. Les délais d'opposition sont différents selon les administrations et le type d'établissement : ainsi, le maire dispose de huit jours, les services de l'État d'un mois pour le premier et le second degré, et de deux mois pour l'enseignement technique. Enfin, et ce n'est pas le moins important, les motifs d'opposition diffèrent selon le type d'établissement : les services de l'État peuvent fonder leur refus sur les motifs tirés de l'hygiène et des bonnes moeurs et, seulement pour l'enseignement technique, de l'ordre public. Le cadre juridique actuel, qui juxtapose donc trois régimes déclaratifs différents du point de vue tant des délais que des motifs d'opposition, est aussi complexe pour les porteurs de projet d'établissement que pour les quatre administrations qui le mettent en oeuvre. oeuvre. Ce régime complexe est aussi incomplet, parce que le cadre juridique actuel ne permet pas de s'opposer à l'ouverture d'une école par un porteur de projet qui aurait été condamné pour des faits graves, par exemple un viol sur mineur. Dans ce cas, l'administration doit attendre que cet individu ouvre son école, puis elle peut déclarer cette illégalité au procureur, qui peut alors saisir le tribunal correctionnel, qui, lui-même, peut condamner l'individu. Entre-temps, des dangers auront été encourus par les élèves. Cette proposition de loi permet de simplifier et d'unifier le régime d'ouverture des établissements hors contrat. Avec les amendements déposés par Mme la sénatrice Françoise Gatel, elle répond à trois objectifs premièrement, simplifier et unifier le régime d'ouverture de tous les établissements hors contrat ; deuxièmement, unifier les délais d'examen des dossiers ; troisièmement, moderniser les motifs d'opposition pour les rendre plus opérants. Je voudrais revenir sur chacun de ces trois éléments. Tout d'abord, pour parvenir à un régime plus simple, les trois régimes actuels seraient remplacés par un régime unique de droit commun. Le cadre juridique actuel prévoit en effet une double saisine, celle du maire, puis celle des trois représentants de l'État. Cette double saisine est source d'insécurité juridique, tant pour les administrations chargées d'instruire les dossiers que pour les déclarants.

puisque les motifs d'opposition seraient unifiés et modernisés. La notion générale d'ordre public, déjà utilisée aujourd'hui pour le seul enseignement technique, serait généralisée à tous les degrés de l'enseignement, les notions plus anciennes étant actualisées par la référence à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Par ailleurs, les motifs permettant d'ores et déjà de demander la fermeture d'un établissement- absence de diplôme du directeur, condamnation pour crime ou délit contraire aux bonnes moeurs -pourraient désormais être opposés à l'ouverture des établissements. La proposition de Mme la sénatrice Françoise Gatel de rendre obligatoire le contrôle des établissements privés hors contrat lors de la première année de leur fonctionnement me semble donc absolument justifiée. Je m'y engage devant vous : le ministère de l'éducation nationale se donnera les moyens, notamment dans les académies où se concentrent les ouvertures de tels établissements, de rendre ce contrôle systématique dans la première année de fonctionnement d'un nouvel établissement. C'est pourquoi cette proposition de loi aura un impact potentiel sur l'organisation de l'éducation nationale, qui doit s'adapter à ces réalités nouvelles. Ces contrôles seront réalisés en étroite collaboration avec l'ensemble des services de l'État, au premier rang desquels le ministère de l'intérieur, lequel dispose d'informations parfois utiles pour prévenir des ouvertures qui ne seraient pas souhaitables. Enfin, troisième et dernier point, qui est extrêmement important, cette proposition de loi permet de trouver un juste équilibre entre liberté d'enseignement et protection des enfants.

Je suis donc extrêmement attentif à ce qu'il n'y soit pas porté atteinte. Je ne vous cache pas que les qualificatifs rappelés par Mme la sénatrice Françoise Gatel m'ont paru tout à fait désobligeants par rapport à l'objectif visé. visé. En réalité, il est question, au travers de cette proposition de loi, de conforter la liberté d'enseignement, en évitant, comme pour toute liberté, que l'abus de cette liberté ne vienne abîmer cette liberté. Toute liberté, Toute liberté, en effet, peut comporter des abus. C'est en étant soigneux vis-à-vis de ces abus que l'on est soigneux vis-à-vis de ces libertés. Je peux vous témoigner de l'intérêt que je porte à toutes les pédagogies alternatives. À cet égard, je suis extrêmement attentif à ce que l'école publique soit elle-même porteuse de ces pédagogies alternatives.

En tant que ministre de l'éducation nationale, je me dois de garantir la protection des enfants et le respect des valeurs de la République dans toutes les écoles en France. La liberté d'enseignement, comme toutes les libertés, pour demeurer, doit s'accompagner d'un cadre clair, partagé et respecté par tous les acteurs. Les valeurs de la République sont le socle de notre action. Lorsque l'école ne porte pas ces valeurs, elle ne se porte plus, et c'est notre société qui en pâtit. Oui, c'est en menant un combat commun pour réaffirmer les valeurs républicaines que nous pourrons renforcer la liberté de l'enseignement. C'est un sujet qui doit unir l'ensemble de la représentation nationale : c'est en dénonçant ensemble ceux qui s'abritent derrière la liberté de l'enseignement pour bafouer les valeurs de la République que nous consoliderons cette Cette proposition de loi permet de définir le cadre nécessaire et attendu au service de la liberté de l'enseignement et de la République. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, comme son nom l'indique, la présente proposition de loi tend à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. C'est pourquoi il me semble important de le dire, et de le répéter à ceux qui s'en inquiéteraient : il n'est nullement question ici d'empêcher l'ouverture d'écoles privées, et encore moins de porter atteinte à une promesse républicaine qui nous est chère, celle de l'école libre. Notre rôle de parlementaires est d'y veiller et de rassurer ceux qui expriment leurs craintes à ce sujet. L'objet de ce texte est en réalité très simple. Il tend à moderniser le régime juridique complexe et dépassé encadrant l'ouverture de ces établissements et apporter ainsi une réponse au vide laissé par la censure du Conseil constitutionnel. Je salue à ce titre l'initiative courageuse de notre collègue Françoise Gatel qui, en reprenant une disposition adoptée ici même lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, propose une solution dans un débat que nous savons très délicat. Par-delà les passions qu'il déchaîne, ce débat est d'abord né de constats que nous partageons sur toutes ces travées. D'abord, il s'agit d'un phénomène bien réel. Le rythme d'ouverture des établissements hors contrat atteint quelques dizaines par an, avec une accélération du nombre de demandes dans le premier degré : le nombre d'écoles et d'élèves y a plus que doublé entre 2011 et 2017. Ensuite, le régime juridique encadrant l'ouverture des écoles privées Aujourd'hui, ces établissements peuvent être ouverts très facilement, chacun le sait, sur simple déclaration, pourvu que soient remplies quelques conditions somme toute basiques. Le droit n'offre donc qu'un régime d'opposition inopérant avec un délai de huit jours pour le maire et d'un mois pour l'État. La réalité que nous vivons a dépassé le droit en vigueur et laisse bien souvent élus et recteurs devant le fait accompli, totalement désemparés. Enfin, les déviances recensées dans certains établissements sont, elles aussi, bien réelles. Nous avons parlé de radicalisation religieuse, de sectarisme, voire d'indigence pédagogique. Je considère qu'il n'est pas utile de pointer du doigt tel ou tel type d'établissements. À mon sens, cela révèle avant tout l'inadéquation du droit actuel face à ces situations. Aussi exceptionnelles soient-elles, elles existent bel et bien et mettent tous les enfants en danger. Nous ne saurions, au nom d'une liberté, en être complices par notre inaction ; je crois, là encore, que nous en sommes tous conscients. Mes chers collègues, en partageant ce diagnostic, nous reconnaissons de fait la diversité de ces écoles, leur nombre, mais aussi la nécessité de rénover un cadre juridique vieux d'un siècle. Je regrette que nos débats en commission ne l'aient pas mis en évidence. Dans le même temps, je pense que ces divergences étaient nécessaires pour prendre le temps de la réflexion et être capables aujourd'hui de replacer non pas l'église, mais la mairie, au centre du village. Je comprends la frustration de ceux qui pensent que ce texte ne va pas assez loin, qu'un régime d'autorisation préalable lui serait préférable. N'y a-t-il pas pourtant une différence, en matière d'exercice d'une liberté fondamentale, entre une déclaration à l'administration et la demande d'une permission ? Mes chers collègues, il s'agit bien de déterminer les conditions d'exercice d'une liberté fondamentale. Notre groupe reste donc attaché à l'idée d'un régime déclaratif renforcé qui trouve un point d'équilibre au sein même de cette liberté d'enseignement que nous chérissons tous, entre le droit de créer une école privée et le droit des parents à choisir l'instruction de leur enfant. Là où nous le placerons, le curseur déterminera non pas notre degré d'attachement à l'école républicaine, mais notre niveau de responsabilité pour assurer à la fois la protection des enfants et la possibilité d'ouvrir un établissement. De même, certains de nos collègues ont évoqué en commission le cas des enfants déscolarisés ou accueillis dans des structures déclarées ou non. J'attire leur attention sur la mise en garde pertinente de notre rapporteur. Là encore, placer la barre trop haut risquerait, nous le savons tous, de reporter une partie des projets d'école vers l'instruction à domicile et les écoles clandestines. C'est pourquoi il nous faut avoir un discours clair vis-à-vis des écoles privées hors contrat il n'est pas question d'empêcher leur création. S'il nous faut permettre aux enfants l'accès à l'enseignement dispensé dans ces établissements, il est indispensable de les maintenir dans un cadre déclaré et contrôlé. Pour ces raisons, nous sommes favorables à ce que ce régime déclaratif évolue vers un dispositif plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées. Ce texte prévoit par ailleurs de mieux contrôler les écoles privées hors contrat. Si un contrôle annuel semble difficilement réalisable, il est impératif de renforcer les contrôles inopinés. Je suis donc favorable à ce que les inspections prescrites lors de la première et de la cinquième année de fonctionnement non seulement deviennent obligatoires, mais qu'elles soient complétées par un contrôle supplémentaire lors de la troisième année. s'agissant des enseignants, nous devons pouvoir procéder aux vérifications de moralité nécessaires, qui sont déjà réalisées pour leurs homologues du privé sous contrat et de l'enseignement public. Mes chers collègues, nous allons maintenant débattre de ce texte en défendant ardemment nos convictions respectives. Je pense néanmoins que personne ici ne peut se satisfaire du. Il est de notre responsabilité de prendre toutes les précautions nécessaires et d'assurer notre rôle de garants des libertés. J'espère donc que nous saurons trouver ensemble une solution

Merci Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a suscité des passions irrationnelles et des oppositions violentes qui ne se sont pas toujours développées dans des formes très démocratiques. C'est regrettable Il est grand temps de revenir à l'essentiel, au droit, et j'espère que notre débat contribuera à une appréhension plus rationnelle de la situation des établissements d'enseignement hors contrat. Une discussion sur le fond aura l'avantage de nous imposer le respect de la laïcité et donc de ne pas juger les motivations pédagogiques, philosophiques ou religieuses des personnes ou des organismes qui souhaitent ouvrir, hors contrat, des établissements d'enseignement. La Constitution reconnaît la liberté d'enseignement, mais ce droit ne s'exerce pas en dehors de tout cadre légal. Je pourrais résumer ce principe en disant que la liberté de circulation n'empêche pas le code de la route. treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantit « l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». L'obligation d'instruction se réalise donc selon des normes générales que la loi définit assez précisément. L'article L. 131-1-1 du code de l'éducation dispose ainsi : « Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté Cette obligation d'une instruction répondant à des principes généraux s'applique aussi dans le cadre familial, quand les parents décident d'organiser eux-mêmes l'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. Un décret de 2012 en a précisé les modalités. Dans le même esprit, pour les établissements hors contrat, le décret du 28 octobre 2016 a défini les compétences attendues des élèves et la manière dont elles sont évaluées. L'article R. 131-13 du code de l'éducation précise ainsi : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire À la suite d'un recours, ce décret a été examiné et validé par le Conseil d'État. Il ne faudrait pas que la loi votée par notre assemblée abolisse ou atténue la portée de ces dispositions de bon sens. De même, notre travail législatif serait préjudiciable s'il avait pour conséquence d'intégrer dans le domaine de la loi des dispositions qui, aujourd'hui, relèvent de la réglementation. La sécurité juridique n'impose pas d'encombrer la loi de dispositions relevant de normes inférieures, bien au contraire. Restons donc dans le cas particulier du régime d'ouverture des établissements hors contrat, qui dépend, cela a été dit, de textes anciens et d'application difficile, notamment pour les maires qui doivent gérer, sans outil juridique efficace, des situations parfois complexes. Légiférons donc, chers collègues, avec le double objectif de leur être utiles et de ne pas mettre à bas l'ensemble des dispositifs qui assurent déjà le contrôle de ces établissements. Ce fut le dessein d'un cavalier législatif justement sanctionné par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 26 janvier 2017, sur la seule base de l'article 38 de la Constitution, celui-ci refusant d'examiner, sur le fond, les griefs des requérants. L'imperfection juridique demeurant, la présente proposition de loi tente d'y apporter une solution, et je porte au crédit de Mmes Françoise Gatel et Annick Billon d'avoir poursuivi initialement ce seul but. Le texte qui nous est proposé, dans sa version amendée par notre commission, est le résultat d'un compromis qui tente de concilier la nécessité d'un contrôle renforcé et la défense du droit à l'enseignement qui va au-delà de ce que les textes garantissent déjà de façon satisfaisante et en conformité avec nos principes constitutionnels. Comme tout compromis, il ne satisfera pleinement personne, et je crains que le régime déclaratif qu'il propose ne s'avère, à l'usage, pas aussi efficient que les acteurs du terrain auraient pu le souhaiter. Je continue de penser que l'avantage d'autoriser un établissement, quel qu'il soit, est justement de pouvoir lui retirer cette autorisation en fonction de règles connues et d'observations clairement établies et contestables devant les juridictions administratives. Au-delà de ce problème de droit restera entière la question des moyens. Contre les opérations d'endoctrinement, les conditions d'enseignement indignes et les risques de sévices, la seule politique efficace consiste à renforcer considérablement les capacités d'inspection de ces établissements par les services de l'éducation nationale. Sur ce point précis, monsieur le ministre, nous attendons de votre part des engagements fermes sans lesquels le dispositif que nous allons instituer par la loi, quelle que soit sa nature, sera inopérant. Je vous remercie Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, les sénateurs du groupe Union Centriste ont souhaité l'inscription à notre ordre du jour d'une proposition de loi visant à simplifier et à mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat. Il faut tout d'abord rappeler qu'il existe actuellement environ 1 300 établissements scolaires hors contrat pour un peu moins de 8 000 établissements sous contrat. Mais, et cela est très inquiétant, le rythme d'ouverture d'établissements hors contrat, de quelques dizaines par an, est en forte augmentation, cela a été rappelé tout à l'heure, en particulier dans le premier degré. les services de l'État reçoivent des signalements de plus en plus nombreux à l'encontre d'établissements dans lesquels le contenu de l'instruction serait très faible ou d'établissements dont l'enseignement ne correspondrait pas aux valeurs de la République. Des dérives sont constatées : Mme la rapporteur a ainsi parlé de « phénomènes de radicalisation pédagogique, de sectarisme, d'amateurisme ou d'insuffisance pédagogique Des dérives inquiétantes, les dangers que représentent certains établissements, la faiblesse, voire la dangerosité de la pédagogie suivie, tout cela n'est pas nouveau et n'avait pas échappé au gouvernement précédent. Ainsi, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, le président de notre groupe Patrick Kanner, alors ministre, avait défendu, au nom du Gouvernement, une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance pour revoir le régime déclaratif d'ouverture des établissements privés hors contrat afin de l'aligner sur le régime d'autorisation préalable actuellement en vigueur en Alsace-Moselle. Au nom de la liberté d'enseignement, l'auteur de la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui s'était, à l'époque, vigoureusement opposée à la proposition du ministre et avait fait voter par la majorité sénatoriale- la même la même qu'aujourd'hui ... -une révision du régime déclaratif d'ouverture. La suite, chacun la connaît : l'Assemblée nationale avait préféré rétablir son texte initial qui fut censuré par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme ... Ah ! ... contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs du présent texte. Aujourd'hui, dans sa proposition de loi initiale, notre collègue Françoise Gatel reprend globalement le texte de l'amendement qu'elle avait fait adopter en 2016. La seule nouveauté réside à l'article 3 il s'agit du renforcement des conditions requises pour diriger ou enseigner dans un établissement privé du second degré. Pour nous, sénateurs socialistes, il paraît toujours et plus que jamais nécessaire de modifier le régime obsolète d'ouverture des établissements privés hors contrat pour pouvoir mettre fin aux dérives précitées constatées. aux dérives précitées constatées. C'est un sujet sensible et complexe, soumis à des influences opposées, parfois virulentes, et l'équilibre entre toutes les contraintes juridiques est difficile à trouver. Nous tenons à souligner que nous ne portons pas de jugement à l'encontre de l'enseignement privé sous contrat, qui, lui, joue globalement bien son rôle dans le respect des règles fixées. En revanche, nous sommes inquiets du développement foisonnant des écoles hors contrat, des établissements qui prolifèrent sous le régime peu regardant de la simple déclaration actuellement en vigueur. À la lecture du texte de cette proposition de loi, il nous est apparu d'emblée qu'il existe un décalage entre l'objectif annoncé, qui montre une prise de conscience des risques de la part des rédacteurs du texte, et la réalité du dispositif proposé qui nous paraît beaucoup moins ambitieux dans son application. L'article 1se contente de renforcer le régime de déclaration d'ouverture des établissements privés hors contrat. Oui ! Là où un régime d'autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l'éducation et à une instruction porteuse des valeurs de la République,

Ce dispositif présenterait une garantie bien supérieure à celle de la simple déclaration, quand bien même celle-ci serait assortie de contrôles plus nombreux et plus systématiques. Une Une procédure d'autorisation préalable à toute ouverture nous paraît aussi largement préférable, car, après l'ouverture d'une école, si cette dernière pose problème, les possibilités d'action de l'État et des élus sont réduites avec le système de la déclaration : chacun est mis devant le fait accompli

Passer à un régime d'autorisation ne serait pas attentatoire à la liberté d'enseignement ni à celle d'association, et encore moins au libre choix d'éducation des familles, puisque cette procédure existe déjà dans notre pays actuellement, en Alsace-Moselle,

On constate par ailleurs que la proposition de loi crée un régime unique d'ouverture d'établissement scolaire privé, mais s'avère « moins-disante » que le texte existant en termes de capacité et de compétence demandées à la personne souhaitant ouvrir un tel établissement., nous pensons qu'il convient de s'aligner sur le contenu des déclarations d'ouverture le plus complet, soit celui des établissements du second degré général contenu dans l'article L. 441-5 en vigueur. Ce sera l'objet de notre deuxième amendement sur l'article 1. Par ailleurs, dans le souci de protection de l'intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, et en référence à l'article 706-47-4 du code pénal, il convient de mentionner explicitement l'interdiction, pour toute personne signalée à l'administration pour des antécédents judiciaires, de tout lien avec un établissement d'enseignement. est l'objet de notre troisième amendement qui vise à créer un article additionnel après l'article 1. Pour ce qui concerne l'article 2 de la proposition de loi, nous souhaitons soutenir l'amendement que Mme la rapporteur Annick Billon

la première, bien entendu, pour contrôler que les choses se passent bien ; la troisième, parce que l'on est en milieu de mandat ; et la cinquième, parce que c'est le moment où l'école privée hors contrat peut demander à passer sous le régime du contrat. Nous souhaitons aussi harmoniser les conditions d'exercice prévues pour diriger un établissement scolaire privé hors contrat en exigeant au moins la même expérience pour le premier et second degré. Actuellement, vous le savez, mes chers collègues, aucune expérience professionnelle n'est exigée pour le premier degré-

de sectarisme, d'amateurisme, voire d'insuffisance pédagogique » qui règnent actuellement dans l'ouverture de ces écoles privées hors contrat. Vous avez cité des abus et des cas qui montrent la difficulté de fermer ou d'empêcher l'ouverture de certains établissements où les enfants seraient en danger. Il ne suffit pas de constater, de regretter ou de se plaindre. Il convient d'agir et de protéger notre jeunesse de ces risques que nous avons évalués et que nous voulons, tous ici, combattre. Reconnaissez-le, il serait regrettable que, après un tel débat entre nous et en toute connaissance de cause des risques encourus, on puisse continuer à ouvrir une école plus aisément qu'un bar ou un restaurant Certes, les dispositions de votre proposition de loi constituent une avancée, ... Ah, quand même ! ... mais nous vous proposons d'aller plus loin, en particulier en soumettant à autorisation l'ouverture des établissements privés hors contrat et en renforçant réellement l'efficacité des contrôles. La parole est à M.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi relative à l'encadrement des établissements privés hors contrat. Ces derniers sont aujourd'hui 1 300 sur le territoire national, dont 300 établissements confessionnels. Notre assemblée doit respecter la liberté d'enseignement, mais elle doit aussi légiférer pour établir des règles strictes en matière d'ouverture et de contrôle de ces écoles. Notre groupe a d'ailleurs déposé un amendement tendant à changer le titre de cette proposition de loi- amendement soutenu à l'unanimité en commission -pour insister sur la nécessité de continuer, année après année, à observer scrupuleusement ces établissements. s'ils sont autonomes financièrement, ces établissements disposent aussi d'une liberté dans l'application des programmes scolaires ou de la méthodologie pédagogique. Tout en célébrant cette liberté, n'oublions pas, mes chers collègues, ce que notre système éducatif doit à notre histoire. Les lois Ferry sur l'école laïque, gratuite et obligatoire, la réforme Berthoin sur l'allongement de la scolarité, la modernisation de l'enseignement à la suite du rapport Langevin-Wallon : ces acquis doivent bénéficier à tous, écoles publiques ou privées, sous contrat ou hors contrat.

! À l'heure de la désinformation et dans un contexte de radicalisation de certaines écoles, il est nécessaire que le Gouvernement, d'un côté, et les services municipaux, de l'autre, puissent rapidement intervenir pour empêcher l'ouverture d'une école contraire aux valeurs de la République. Cette proposition de loi tend à donner des moyens efficaces aux acteurs nationaux et aux acteurs locaux : allongement des délais d'opposition, uniformisation des motifs d'opposition, contrôle annuel des établissements et nouvelles conditions à l'enseignement dans ces établissements hors contrat. Des situations comme celle récemment rencontrée à Toulouse ne sont pas tolérables en France. La République ne saurait subir un tel affront. Après des années, après des siècles de lutte contre l'obscurantisme, pour l'éducation universelle et l'accès libre à la connaissance, notre parlement doit protéger ces acquis par tous les moyens nécessaires. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants est très sensible à cette proposition de loi et présentera une série d'amendements pour l'enrichir. L'éducation est un droit durement acquis : sachons le préserver en établissant un équilibre précis entre liberté de l'enseignement, rigueur scientifique et respect des valeurs républicaines. La parole

Les écoles privées hors contrat ont prouvé, par leur diversité et leurs spécificités, qu'elles occupaient une place bien particulière dans l'offre éducative française. Alors, nous sommes en droit de nous, de vous poser la question : pourquoi pourquoi s'attaquer aux écoles indépendantes, elles qui ne représentent qu'une part infime d'élèves ? Elles accueillent 70 000 enfants sur les 12 millions d'enfants scolarisés en France. Ces écoles proposent des schémas divers et variés utilisant des méthodes d'enseignement et de pédagogie qui doivent être préservées et regardées de près. car elles sont le fruit d'une liberté constitutionnelle d'enseigner ; regardées de près, car le succès de ces écoles doit nous interpeller face aux grandes difficultés de l'éducation dite « nationale Alors même que le Conseil constitutionnel avait censuré la disposition créant un régime d'autorisation préalable pour l'ouverture d'écoles hors contrat, disposition décidée par la non regrettée Mme Vallaud-Belkacem ... Un peu de respect ! ... dans le projet de loi Égalité et citoyenneté, vous revenez à la charge, car cette proposition revient à faire subir les mêmes conséquences. C'est très pernicieux. Votre démarche est en réalité insincère et cache mal votre volonté d'entraver une liberté pourtant fondamentale. Rappelons que le Conseil constitutionnel avait rejeté le régime d'autorisation préalable, parce qu'il « portait une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d'enseignement, indissociable de la liberté d'association Les conditions drastiques que pose votre proposition sont beaucoup trop contraignantes et seront, n'en doutons pas, un frein considérable à l'ouverture d'écoles indépendantes. Je crains que ce ne soit là votre but inavoué. Sous couvert de bons sentiments, et notamment d'une urgence absolue, que nous soutenons, de lutte contre l'islamisme radical, on en vient à soupçonner, voire à punir tout le monde, et finalement toutes les écoles indépendantes, dont un certain nombre sont chrétiennes, et qui, elles, n'ont rien à se reprocher. Ne serait-ce pas votre but, mes chers collègues ? Si cela ne l'était pas directement pour tous, les ayatollahs de la laïcité et les adversaires de notre modèle républicain reposant sur la liberté, et notamment sur la liberté d'enseigner, se frottent déjà les mains. concerne la volonté plus que légitime de surveiller les écoles quant aux risques de transmission d'un islam radical, il conviendrait de développer les contrôles en aval. C'est une hypocrisie totale de s'attaquer aux écoles hors contrat, ... Ah ! ... alors que l'islam radical se propage dans la clandestinité, le plus souvent lors de cours

permettez-moi de préciser que, au titre du dernier projet de loi de finances, aucun poste n'a été attribué à l'enseignement privé sous contrat, alors que, depuis les accords de 1992, l'État s'était l'État s'était engagé à respecter la règle des 80-20 : 80 % de postes pour le public et 20 % pour le privé. Pour conclure, je tiens à dire que l'ensemble de ces éléments nous poussent à croire que le Gouvernement cherche à briser l'essor des écoles hors contrat, alors qu'il est de sa responsabilité aimons la liberté ! Je le dis clairement : le Front national est intrinsèquement pour la liberté d'enseignement, car c'est une liberté fondamentale. Nous devons la chérir et non la flétrir.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans le, plus précisément à l'article consacré à la liberté de l'enseignement, le radical Ferdinand Buisson écrivait : Mais de ce que nul citoyen, dans un pays libre, ne peut être arbitrairement privé du pouvoir d'enseigner, s'ensuit-il que ce pouvoir soit en quelque sorte un droit de nature, illimité, inconditionnel, et dont l'exercice ne soit subordonné à aucune règle, à aucun contrôle ? Pour répondre à cette question, il suffit de se demander s'il s'agit là d'un droit dont l'exercice intéresse l'individu seul. N'est-ce pas évidemment au contraire un droit qui s'exerce à l'égard de mineurs, c'est-à-dire de personnes dont l'État est le protecteur naturel ? » Tout à fait ! Le groupe du RDSE fait sienne cette conception de cette liberté et refuse que l'on puisse tolérer d'« abuser impunément de la faiblesse de l'enfance Comme pour toute liberté, son exercice a pour limite le droit d'autrui : en l'espèce, le droit de l'enfant à l'instruction consacré par le préambule de la Constitution et par la convention européenne des droits de l'homme. Il ressort d'ailleurs de la jurisprudence européenne que l'État est responsable des écoles publiques et privées ; qu'il a pour obligation de sécuriser ce droit et de protéger les élèves contre les mauvais traitements au sein des écoles. La République a donc la responsabilité de prévenir toute dérive. Elle doit garantir un droit à l'instruction, dont tous les enfants ne semblent pas bénéficier, malheureusement, même s'il s'agit d'une infime minorité. D'ailleurs, la circulaire du 17 juillet 2015 relative au régime juridique applicable à l'ouverture et au fonctionnement des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat confirme que l'absence de contrôle peut entraîner la responsabilité de l'État. La liberté de l'enseignement, principe à valeur constitutionnelle, emporte certes des droits, comme celui d'établir un projet pédagogique alternatif ou de percevoir un financement public sous certaines conditions pour les établissements sous contrat, mais elle a toujours comporté des limites, qu'il est loisible au législateur de fixer. Ainsi, les nouvelles conditions d'ouverture des établissements privés hors contrat sont avant tout destinées à vérifier, d'une part, que ceux-ci présentent bien un caractère scolaire et, d'autre part, que le respect de l'ordre public et la protection des enfants accueillis sont assurés. Remettons les choses dans leur contexte : en quoi le fait de constituer un dossier- peu importe sa forme -entraverait-il la liberté d'enseignement, dès lors qu'il s'agit de se prémunir contre des dérives idéologiques ou religieuses non conformes aux valeurs de la République ? J'insiste sur ce point : la proposition de loi ne remet en cause ni le libre choix des parents quant à l'éducation de leurs enfants ni les pédagogies qui peuvent être proposées par ces établissements. Il n'est porté aucune restriction à leur autonomie. Les structures sérieuses que nous connaissons tous n'ont rien à craindre des dispositions proposées. Nous soutenons donc les grandes lignes de cette proposition de loi, bien que notre préférence aille à un régime d'autorisation. Voilà ! L'harmonisation des procédures met fin à une sédimentation incompréhensible. L'actualisation des motifs d'opposition était indispensable, de même que l'allongement des délais d'opposition, notamment pour les maires, pour qui le délai d'examen de huit jours est trop bref. Je tiens également à saluer la mise en place d'un guichet unique. Pour tout dire, nous estimons que cette proposition de loi ne va pas assez loin. Le régime déclaratif n'est pas entièrement satisfaisant. La création d'un régime d'autorisation permettrait de suspendre ou de retirer l'autorisation. Nous tenons à rappeler que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'incompatibilité d'un tel régime avec la liberté d'enseignement. En outre, il est essentiel de faciliter la détection d'éventuelles maltraitances et agressions sexuelles. À ce titre, exiger le bulletin n° 2 du casier judiciaire, lors de la constitution du dossier, à l'instar de ce qui se fait pour les enseignants du public et du privé sous contrat,

C'est le sens de l'un de nos amendements et de plusieurs sous-amendements que nous défendrons. En la matière, le droit en vigueur est insuffisant. Par ailleurs, l'amende de 15 000 euros en cas de non-respect des conditions d'ouverture n'a qu'une faible portée dissuasive au regard des sommes dégagées par certains établissements. Je regrette enfin le sort réservé à notre amendement tendant à instaurer un contrôle médical des élèves scolarisés dans les établissements privés hors contrat, frappé par l'article 40 de la Constitution. Proposée par le rapport de la commission d'enquête sur les dérives sectaires, qu'a établi notre ancien collègue Jacques Mézard, cette mesure instaurait une véritable prévention en matière de santé et de protection de l'enfance. Mes chers collègues, nous sommes conscients que l'efficacité de la proposition de loi se mesurera aux moyens d'inspection déployés aux fins de contrôle. Le fait de prévoir que celui-ci s'exerce obligatoirement lors de la première année risque toutefois de fausser l'image que l'on peut avoir de l'établissement. Le nombre de contrôles a certes été renforcé. J'espère que le Gouvernement pourra nous éclairer quant aux actions qu'il compte entreprendre pour améliorer la réactivité de l'État face aux dangers réels auxquels sont exposés certains enfants.

de manifestations et de contestations entre les tenants de ce principe et les partisans de la seule école publique. Le projet de loi du ministre Alain Savary a été l'un des moments forts de ces affrontements. Le 24 juin 1984, deux millions de personnes ont défilé dans les rues de Paris pour signifier leur opposition à ce projet, contraignant le Président François Mitterrand à faire marche arrière. La moindre étincelle rallume l'incendie. J'ai pu le constater, en 2009, lors des débats sur ma proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Si ce texte a permis de résoudre la quasi-totalité des situations qui enflammaient l'ordre du jour du congrès des maires, je suis toujours épinglé au tableau noir de certaines organisations, qui considèrent que l'argent du contribuable doit être strictement réservé à l'école publique. Plus récemment, le précédent gouvernement, dans le texte Égalité et citoyenneté, a voulu substituer au régime de déclaration d'ouverture des écoles privées un régime d'autorisation. Le Conseil constitutionnel, que nous avions saisi, a annulé le dispositif, qui recourait aux ordonnances. Aujourd'hui, la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel vise à faire face à une situation nouvelle : le risque de radicalisation. Ce texte conserve le dispositif de déclaration et préserve la liberté d'enseignement, à laquelle nous la savons attachée. Bien entendu, cette liberté, comme toutes les libertés, doit être « encadrée », notamment lorsque la sécurité est en jeu. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. liberté. Mes chers collègues, il est de notre devoir d'assurer la sécurité physique, morale et sanitaire de tous les élèves et des personnels de la communauté éducative

Si le phénomène de radicalisation est récent, l'école a toujours été l'enjeu de mouvements sectaires. Cette situation avait conduit, en 1998, Mme Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l'enseignement scolaire, à adapter le cadre législatif existant en soutenant deux propositions de loi sénatoriales, dont j'ai été le rapporteur, qui renforçaient le contrôle de l'obligation scolaire. Aujourd'hui, même si ce risque est limité, nous devons tout mettre en oeuvre pour lutter contre la radicalisation. Dans le même temps- si vous me permettez cette expression -, nous ne devons pas porter atteinte aux établissements qui, en optant pour le hors contrat, choisissent des méthodes et des pédagogies différentes donnant de bons résultats, ce à l'heure où notre école publique envoie au collège 30 % d'enfants qui ne savent pas suffisamment lire, écrire et compter. Or l'éducation nationale et, d'une manière plus large, l'administration sont souvent pointilleuses, sourcilleuses, voire rétives à certaines innovations ou expérimentations. De ce fait, elles ont souvent une interprétation

Ces raisons nous conduisent à approuver la proposition de Françoise Gatel, rapportée par Annick Billon, de fixer dans la loi une liste des pièces déclaratives ; c'était l'objet de plusieurs de nos amendements, que nous avons retirés en commission au profit des amendements identiques de Mme Gatel. s'agit d'une liberté constitutionnelle, et le diable se cachant souvent dans les détails, c'est au législateur de définir les critères d'appréciation et non à une juridiction par voie de décret. Je tiens à saluer le travail accompli par notre rapporteur. Sur un sujet passionnel, elle a su conforter la proposition de Françoise Gatel. Mme le rapporteur vient de détailler les mesures en question ; mes collègues y reviendront s'ils le souhaitent. Permettez-moi, pour ma part, de retenir quelques avancées : l'uniformisation des délais, le guichet unique et le renforcement des contrôles. C'est en effet au cours ou au terme de la première année que les risques seront visibles. Au moment de la déclaration, les demandeurs dont nous redoutons les projets seront suffisamment habiles pour masquer leurs intentions. J'y reviendrai lors de la discussion de notre amendement visant à associer à ces contrôles, sous l'autorité du préfet, les services compétents du ministère de l'intérieur. collègues, vous l'aurez compris, notre groupe, attaché à la liberté fondamentale du libre choix de l'école, votera cette proposition de loi de Françoise Gatel, rapportée par Annick Billon, parce qu'elle conjugue liberté et sécurité. La parole

À ce titre, ces enfants ont le droit d'étudier dans des conditions d'accompagnement pédagogique et de sécurité satisfaisantes. Face à la radicalisation croissante de certains établissements ou face au risque d'indigence éducative, face au danger potentiel qui en résulte pour les élèves, cette proposition de loi apporte des solutions pour traiter plus efficacement les situations les plus inquiétantes et éviter le développement de nouvelles dérives.

d'abord, la procédure est complexe et source d'ambiguïté. Ensuite, les moyens d'action sont limités, et l'impossibilité d'agir pour les élus locaux et les services de l'État amène à ce qu'ils soient souvent placés devant le fait accompli. Malgré l'évidence de situations identifiées comme graves, les procédures ne répondent pas à l'urgence. Ce qui frappe, c'est qu'il y a aujourd'hui une incohérence entre, d'un côté, la capacité dont dispose l'État à agir rapidement et fermement dans les établissements publics ou privés sous contrat, d'ailleurs parfois sur injonction des parents ou des enseignants, et, de l'autre, le sentiment de secret et de silence, source de fantasmes plus ou moins fondés, qui peut régner autour des écoles hors contrat. Cette proposition de loi entend donc simplifier et harmoniser les procédures, mieux encadrer et renforcer le régime de déclaration et introduire la transparence nécessaire à la protection des enfants. La proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel intervient dans un contexte où l'enseignement privé hors contrat connaît un véritable essor. Notre rapporteur, Annick Billon, a rappelé les chiffres ; ils sont éloquents. Il y avait 800 établissements scolaires privés hors contrat en 2010. Il y en a aujourd'hui 1 300 ; ils ont donc connu une croissance de plus de 60 %. Ce qui frappe, c'est que 57 % des effectifs concernent le primaire, donc l'entrée des enfants dans la scolarité. Cela signifie un nombre croissant de parents qui choisissent dès le début une école hors contrat pour éduquer leurs enfants. cette question interpelle, bien sûr, même si elle n'est pas l'objet du présent texte, quant aux motivations, quant aux raisons de ce choix délibéré. Elles sont multiples, obéissent certainement à des ressorts différents, mais suscitent toutes une analyse approfondie pour faire évoluer notre propre système scolaire. Je ferme ici cette parenthèse, pour revenir à notre sujet. Aujourd'hui que se passe-t-il ? Quand ces établissements ouvrent, les autorités sont démunies, car l'effectivité du contrôle des établissements est limitée, d'une part, par la brièveté et la disparité des délais d'opposition et, d'autre part, par la restriction des motifs pouvant être invoqués à l'appui d'un refus d'ouverture. rien d'étonnant à tout cela : le régime déclaratif actuel se décline en trois procédures qui datent de la fin du XIX et du début du XX siècle et qui répondent donc à une situation scolaire désormais datée. Il est évident que ce système est devenu obsolète et qu'il doit être réformé. J'y insiste, si ce changement doit s'effectuer, c'est sans porter atteinte à la liberté de l'enseignement. Pourtant, il est indispensable de contrôler ces établissements, faire entrer le regard extérieur de la puissance publique, garante de la neutralité de la République et de la protection des enfants. Tout l'enjeu de cet équilibre est de rendre effectif le contrôle et de préserver la liberté fondamentale de l'enseignement. Cet équilibre est le fondement du présent texte.

La proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel conserve cet équilibre, au travers d'une procédure de déclaration, tout en permettant que des contrôles réels soient effectués. C'est une proposition de loi pragmatique, simplificatrice, dont le but unique est de garantir davantage d'efficience et d'efficacité.

Elle allonge également les délais de recours, uniformise et actualise les motifs de refus d'ouverture et rend plus effectifs les contrôles. En effet, en l'état actuel du droit, le maire ne peut s'opposer à l'ouverture d'un établissement que sur le fondement des « bonnes moeurs »- des bonnes moeurs ? de l'hygiène et des exigences de sécurité et d'accessibilité ». La proposition de loi fixe quatre motifs de refus d'ouverture invocables par le maire, le recteur, le préfet et le procureur de la République. Elle renforce le pouvoir des maires, en leur permettant de s'opposer à l'ouverture pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux. Elle permet également aux services de l'État d'intervenir en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants.

Mes chers collègues, rien n'est plus normal que de demander aux écoles hors contrat de se conformer aux obligations de sécurité et d'accessibilité qui s'imposent à tous les établissements recevant du public. Rien n'est plus normal que d'autoriser la fermeture d'un établissement qui n'a pas le caractère d'un établissement scolaire. Absolument ! Rien n'est plus normal que de renforcer le principe d'un contrôle des établissements hors contrat. Il n'y a rien de liberticide dans tout cela, contrairement au mauvais procès qui a pu être fait à ce texte. Ce qui serait liberticide, ce serait de ne pas fixer un cadre efficace. est un texte de bon sens et d'équilibre. La liberté d'enseigner n'est pas la liberté de tout faire et dans n'importe quelles conditions. Les membres du groupe Union Centriste se félicitent des avancées proposées dans ce texte et vous proposent d'adopter une série d'amendements qui tendent à renforcer l'encadrement de l'ouverture des écoles hors contrat. Avec ce texte, on répond à l'exigence des garanties physiques de sécurité, d'hygiène et d'accessibilité des locaux. Avec ce texte, on répond aussi au besoin de garanties éducatives d'acquisition d'un socle de connaissances élémentaires. Avec ce texte, on répond enfin à l'assurance de garanties morales d'ouverture et d'indépendance d'esprit. La République doit ces garanties aux enfants, quand bien même elle ne prendrait pas en charge leur éducation scolaire. Pour ces raisons relevant de l'évidence, nous vous demandons de soutenir cette démarche en votant cette proposition de loi, qui traite avec pragmatisme d'un encadrement nécessaire et juste. C'est un texte au service de la République, au service de la société et, surtout, au service de nos enfants.

le président de notre groupe, Claude Malhuret, a su résumer tout l'enjeu de cette proposition de loi : trouver un équilibre entre respect de la liberté d'enseignement, rigueur scientifique et préservation des valeurs de la République. En effet, nul ne saurait ignorer les fondements de notre nation et nos valeurs les plus essentielles. C'est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité s'investir concrètement dans l'examen de cette proposition de loi. L'esprit des amendements que nous avons déposés sur ce texte peut se résumer en trois grandes idées. Premièrement, les contrôles concernant l'ouverture d'établissements privés hors contrat doivent être renforcés

pour contrôler chaque nouveau recrutement et s'assurer du professionnalisme des personnels recrutés. Deuxièmement, les contrôles doivent être identiquement renforcés, en aggravant les sanctions pour une ouverture en dépit de l'interdiction du ministère de l'éducation nationale, y compris en prévoyant la possibilité d'une peine de prison en cas de récidive, ou encore en associant les services de la mairie aux contrôles réguliers de ces établissements, au regard de leur bonne connaissance du terrain. Nous nous réjouissons d'ailleurs qu'une proposition identique soit portée par notre collègue Françoise Gatel, auteur de cette proposition de loi. Troisièmement, l'administration doit disposer des moyens nécessaires pour faire respecter ses prérogatives. Il est très regrettable que les nombreux dispositifs existants ne soient que peu, voire pas, appliqués, comme cela a été le cas à Toulouse. Le renforcement des moyens d'action du préfet, voté en commission, va ainsi dans le bon sens. Nos amendements visent donc à permettre le recours à un dispositif de prise en charge éducative et sociale des enfants lorsque leurs parents refusent de les scolariser alors même que leur établissement a été fermé pour non-respect des règles en vigueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants salue l'engagement de cette proposition de loi visant à préserver les valeurs de l'éducation républicaine. Ce texte offre un juste équilibre entre encadrement de l'ouverture et du contrôle des établissements privés hors contrat et respect de la liberté d'enseignement. Il est en effet nécessaire de respecter l'avis des parents et leur choix d'établissement pour la scolarisation de leurs enfants. Nous étudierons avec attention les amendements de nos collègues, et nous espérons vous convaincre de la pertinence des nôtres. La parole est

pour examiner la proposition de loi déposée par Françoise Gatel, dont notre collègue Annick Billon est rapporteur. Je salue leur engagement et leur travail, ainsi que les valeurs républicaines qui les ont guidées dans leurs démarches.

-, en particulier dans l'enseignement primaire. Cela signifie que les effectifs vont mécaniquement augmenter dans les prochaines années. Deuxième constat : les exigences sont faibles s'agissant de la formation des enseignants et des directeurs, sauf pour l'enseignement professionnel- d'autres orateurs l'ont dit avant moi.

les délais d'opposition qui font suite à la déclaration d'ouverture sont trop courts pour être efficaces : huit jours pour une mairie, quelle que soit sa taille, c'est évidemment bien trop peu pour examiner un dossier.

donné quelques assurances dans votre discours liminaire. Vous avez affirmé que vous alliez vous donner les moyens de contrôler

pour assurer le respect de principes clairs, protecteurs des enfants comme des valeurs républicaines. Il faut évidemment renforcer le suivi et les contrôles, qui sont notoirement défaillants aujourd'hui.

Il est important que des établissements puissent apporter une éducation alternative, recherchée par certains parents, pour les enfants dits « porteurs de handicaps », par ceux qui souhaitent un rythme plus adapté. Cependant, l'État ne doit en aucun cas se trouver devant le fait accompli. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé en conclusion : il s'agit de définir ensemble un cadre clair, clair, partagé et respecté par tous. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter en faveur de ce texte. La parole

même panier. Certains d'entre eux peuvent être de véritables laboratoires de pédagogies innovantes et alternatives, notamment pour des enfants à profil particulier, tels que

en revanche, présentent une face plus sombre et constituent de véritables modèles d'enfermement. C'est en tant que corapporteur de la mission d'information sur l'islam en France, dont le rapport a été rendu en juillet 2016, que j'ai souhaité prendre la parole cet après-midi. Pour mener à bien ce travail, nous avions évidemment procédé à bon nombre d'auditions et nous nous étions notamment intéressés à l'enseignement privé musulman. Apparu au début des années 2000, l'enseignement privé musulman a répondu à une demande grandissante de nombreuses familles qui, en plus d'un enseignement répondant aux normes de l'éducation nationale, souhaitaient qu'un projet éducatif répondant aux critères de l'islam soit dispensé à leurs enfants. Là encore, il serait inopportun d'appréhender de manière identique toutes ces écoles confessionnelles musulmanes hors contrat. Certaines d'entre elles peuvent offrir de vrais modèles d'enseignement et d'ouverture, accueillant même des élèves d'autres religions d'autres, en revanche, sont plus fermées et vivent dans un « entre soi », proposant, par la formation confessionnelle, une vision rigoriste et obtuse de l'islam, tout en ayant l'obligation de respecter le socle commun et minimal de connaissances qui s'impose à tout établissement. C'est bien sûr sur cette partie facultative qu'il convient d'être vigilant, car de jeunes enfants ne peuvent disposer d'un esprit critique et le manifester face à ce qu'on leur indique et seront naturellement plus perméables à ce qu'ils recevront. Au cours des travaux de la mission sénatoriale sur l'islam en France, les représentants du ministère de l'éducation nationale nous ont indiqué- il faut le dire ici -que les rapports d'inspection n'ont pas mis en évidence de dérives particulières dans les établissements confessionnels musulmans, comme la radicalisation ou un rejet des programmes ou des valeurs du socle commun, mais ont relevé que les porteurs de projet manquent souvent de connaissance suffisante des attendus et privilégient des méthodes d'apprentissage fondées sur la répétition ou le par coeur,

que dans le contenu du dossier de déclaration, dont on peut penser qu'il sera souvent, sinon toujours, bien préparé et minutieusement ficelé.

fondamental que ceux-ci puissent certifier que les enseignements prodigués au sein de ces établissements ne servent pas à ancrer une quelconque idéologie. Le manque de moyens de Le manque de moyens de l'inspection de l'éducation nationale a, certes, fréquemment été évoqué, mais si nous ne nous donnons pas ces moyens,

de jeunes enfants en otages de leur savoir dès leur plus tendre enfance, dans le but de les enrôler dans une idéologie qui pourrait être contraire aux valeurs de la République. Faut-il rappeler que les chiffres de la radicalisation sont alarmants ? Nous sommes passés en quatre années de 700 signalements à plus de 19 000 ! Je redis ici qu'il ne s'agit aucunement de freiner le développement des établissements hors contrat, bien au contraire. Ceux d'entre eux qui proposent des pédagogies nouvelles méritent d'être encouragés et soutenus. Il ne s'agit pas plus de stigmatiser les écoles privées hors contrat confessionnelles musulmanes, ... Cher collègue, il va falloir conclure ! ... mais il faut être vigilant vis-à-vis de celles qui pratiquent la fermeture d'esprit et prônent des valeurs contraires à celles de la République. je voterai d'autant plus aisément ce texte que celui-ci garantira que les contrôles seront améliorés et renforcés pour les établissements hors contrat, conformément à un amendement déposé par le groupe Les Républicains. La discussion La discussion générale est close. La commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

Cet article confirme que nous restons dans un régime de déclaration, et non d'autorisation préalable, lequel aurait porté atteinte à la liberté d'enseignement, principe à valeur constitutionnelle. Permettez-moi de m'en féliciter. En revanche, l'allongement des délais d'examen et, éventuellement, d'opposition prévu dans cet article donne lieu à débat. Il faut laisser le temps aux administrations concernées d'appréhender le dossier, sans pour autant que ce délai entrave, dans les faits, le projet d'ouverture ou le retarde d'un an. d'un délai raisonnable de trois mois pourrait répondre à cette double exigence. De même, le renvoi à un décret en Conseil d'État, prévu dans le texte d'origine, pose problème. L'amendement déposé par Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi, et, auparavant, par Jean-Claude Carle et Bruno Retailleau, tendant à présenter dans le corps de la loi plutôt que dans un décret la liste des pièces demandées lors de la déclaration d'ouverture protège la liberté d'enseignement de tout risque de prolifération excessive de contraintes qui réduiraient cette liberté. Exiger trois mois à l'avance, comme le propose le texte initial, la liste des professeurs, leurs titres et les volumes horaires par discipline rendrait particulièrement difficile l'ouverture d'une école et porterait atteinte, de fait, à la liberté d'enseignement. Les amendements approuvés ce matin par la commission tendant à écarter toute référence au projet pédagogique, aux horaires et aux programmes permettent d'éviter le risque de soumettre tout projet d'ouverture à une sorte d'imprimatur pédagogique officiel ou de déclaration préalable pédagogique. Toute liberté peut donner lieu à des abus, ce n'est pas une raison pour la réduire à l'excès. L'article 1 de la proposition de loi ne réalisera donc pleinement ses objectifs- mieux encadrer le régime de déclaration sans remettre en cause la liberté d'enseignement

Tous les enfants ont droit, dans notre pays, à un enseignement construit et de qualité, dans le respect des valeurs de la République. Oui, la liberté de l'enseignement existe- les parents disposent d'un large choix pour scolariser leurs enfants -, mais l'État a le devoir d'organiser l'enseignement public gratuit et laïque, et la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement. C'est au législateur qu'il revient de fixer les limites à cette liberté d'enseignement lorsqu'un établissement contrevient à ces principes, afin de mettre un frein aux dérives de toutes sortes. Car celles-ci existent, nous le savons tous ! L'introduction d'une procédure d'autorisation pour l'ouverture d'une école hors contrat, que propose le groupe socialiste et républicain, remettrait pas en cause la liberté d'enseignement. Ce serait au contraire le moyen d'exercer cette liberté. Un système de contrôle offrirait une garantie bien supérieure à celle de la déclaration et permettrait de mieux prévenir les phénomènes de radicalisation religieuse, de sectarisme, d'amateurisme ou d'insuffisances pédagogiques, qui sont une réalité dans un certain nombre d'établissements. Au cours des contrôles effectués dans ces écoles, les inspecteurs les inspecteurs ont principalement relevé une pauvreté pédagogique, ce qui fragilise le développement des enfants. Cela n'est donc pas compatible avec le code de l'éducation. Rappelons que ces établissements hors contrat ont une gestion totalement autonome : ils embauchent qui ils souhaitent aux postes d'enseignants et ne sont pas tenus de suivre les programmes officiels. Il suffit d'avoir plus de dix-huit ans, d'être titulaire du baccalauréat, de nationalité française et de ne pas avoir été condamné par la justice pour pouvoir ouvrir une école avec une simple déclaration. Alors, oui, les dérives existent, et cette mise en danger des élèves est inacceptable Mes chers collègues, quel est notre rôle en tant que législateur ? Il est de protéger au mieux les élèves, de nous assurer de l'égalité des chances, de garantir le respect des valeurs de la République et des principes d'égalité entre les filles et les garçons, de garantir à toutes et à tous un enseignement pédagogique de qualité et de permettre à tous les enfants d'atteindre le socle commun de connaissances. C'est dans ce sens que va l'amendement du groupe socialiste et républicain. Sachons concilier liberté d'enseignement et protection des enfants ! La parole

qui dispose : « Tout ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire est placé sous la surveillance et la direction des autorités de l'État. [ ...] L'autorisation de l'État est nécessaire : [ ...] pour ouvrir une école ; pour engager un maître dans une école. Toute école peut être fermée par les autorités administratives lorsqu'elle ne se conforme pas aux prescriptions officielles en ce qui concerne l'organisation et le programme.

! Madame Gatel, acceptez l'amendement du groupe socialiste et républicain, et lançons-nous dans cette procédure d'autorisation ! Cela étant, je rassure tout de suite les Alsaciens-Mosellans : le code de l'éducation est très clair, la loi que vous voterez ne s'appliquera pas, et nous continuerons à avoir un système d'autorisation

exiger des conditions drastiques avant l'ouverture d'une école, c'est la juger et, dans de trop nombreuses situations, la condamner avant même qu'elle ait pu, ou su, faire ses preuves. En l'état, les conditions drastiques que pose l'article 1 sont beaucoup trop contraignantes et constitueront, n'en doutons pas, un frein considérable à l'ouverture de ces écoles. De plus, il est beaucoup trop dangereux de laisser à un décret le soin de fixer la liste des pièces constitutives d'un dossier de déclaration, tant les gouvernements successifs pourraient, à leur gré, modifier et durcir encore les critères. Les conditions d'ouverture fixées par l'article 1 vident de leur substance les libertés d'enseignement et d'association, puisqu'elles conduisent à soumette à l'appréciation de l'État et du maire le projet pédagogique, les programmes, les titres des professeurs et jusqu'au volume horaire des cours qui sont dispensés. Une telle évolution est en rupture totale avec l'équilibre même du droit issu de la loi Debré et de la jurisprudence constitutionnelle. La liberté d'enseignement des écoles indépendantes est aussi assurée par le fait que celles-ci ne reçoivent aucun financement public. Le comble serait qu'elles soient autant contrôlées que les écoles sous contrat, qui, elles, en bénéficient ! Cette proposition de loi, si elle devait être adoptée en l'état, aboutirait à ce paradoxe. Enfin, l'allongement des délais des délais d'examen du dossier, associé à l'obligation, déjà en vigueur, de communiquer le plan des locaux, contraindrait les créateurs à louer des locaux vides pendant des mois. L'équilibre financier toujours précaire de ces établissements, qui s'autofinancent, serait gravement menacé. Toutes les propositions allant dans ce sens n'auront pour conséquence que de mettre des bâtons dans les roues des écoles indépendantes. C'est une injustice et une erreur auxquelles je m'opposerai, bien entendu.

pour sécuriser à la fois les porteurs de projet et les autorités concernées. Cet amendement tend donc à distinguer clairement le demandeur et le directeur de l'école. Une personne ne peut cependant diriger l'école ou y enseigner, même si elle l'a créée, que si elle remplit les conditions de qualification et d'expérience particulières qui sont présentées à l'article 3.

l'État. Dans un souci de cohérence, les motifs et les délais d'opposition sont unifiés, et donc rallongés pour tous les acteurs. Une information de l'administration est rendue obligatoire en cas de changement d'identité du représentant légal de l'établissement et surtout de son directeur, afin d'éviter que des requérants aient recours à des hommes de paille pour la seule phase d'ouverture. Enfin, le présent amendement vise à inscrire dans la loi la liste des pièces constitutives du dossier.

Le présent sous-amendement vise à rendre obligatoire un contrôle du casier judiciaire du déclarant au moment du dépôt du dossier, afin de vérifier qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'accueil des mineurs.

La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que les privations par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille peuvent ne pas figurer sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire du candidat.

qui prévoit qu'aucun directeur ou qu'aucun employé de l'établissement ne doit avoir fait l'objet de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs. Cette interdiction est essentielle dans un environnement où des mineurs sont accueillis.

recevant la demande d'ouverture disposera d'un délai de quinze jours pour demander les pièces manquantes. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais plus longs.

Ce sous-amendement a pour objet d'apporter une garantie supplémentaire aux porteurs de projet en soumettant explicitement le processus déclaratif au droit commun prévu par le code des relations entre le public et l'administration, Le constat des pièces manquantes par l'administration se fera par principe dans l'accusé de réception du dossier délivré dès la remise du dossier ou, à défaut, dans un délai de deux semaines.

De plus, l'article L. 114-5 du CRPA prévoit que, si l'administration constate que le dossier est incomplet, son délai de réponse court à compter de la réception des pièces manquantes.

le présent sous-amendement vise à circonscrire explicitement à quinze jours le délai dont disposera l'administration pour signaler que le dossier d'ouverture d'un établissement scolaire privé est incomplet. Enfin, pour parfaire ces garanties offertes aux porteurs de projet d'établissement, le sous-amendement tend à préciser que c'est l'autorité académique qui tient informées les autres autorités disposant de la possibilité de s'opposer à l'ouverture, et ce de manière concomitante à chacune des étapes de ce processus.

et la fermeture de l'établissement ; demain, il pourra de plus interdire à l'intéressé de diriger un établissement ou d'enseigner dans un établissement scolaire, ce qui lui interdira aussi d'ouvrir un tel établissement. La durée de l'interdiction est laissée à l'appréciation du juge en fonction des cas. Considérant qu'il est primordial qu'une personne ayant enfreint une décision administrative ne puisse ouvrir de nouveau un établissement en perpétuant les mêmes délits, je vous invite, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement.

Cela portera à trois mois et demi le délai d'examen des dossiers lorsque ces derniers sont incomplets. Cette disposition constitue néanmoins une garantie que l'examen du dossier ne sera pas retardé par manque d'une pièce. Le projet de loi pour un État

Le sous-amendement n° 42 rectifié présenté par Mme Laborde vise à préciser que les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'accueil de mineurs ne peuvent ouvrir un établissement d'enseignement scolaire. Ce point est satisfait par le droit en vigueur.

uniquement aux administrations. L'article 776 du code de procédure pénale prévoit à cet effet qu'il est délivré aux autorités compétentes lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'ouverture d'une école privée.

Cet amendement vise à créer un guichet unique, avec un droit d'opposition pour chacune des quatre autorités administratives aujourd'hui compétentes : le maire, le préfet, le procureur de la République et l'autorité académique. Aucun motif d'opposition nouveau n'est créé. Ceux qui existent aujourd'hui sont étendus à tous les degrés d'enseignement.

objet de renforcer les sanctions encourues en cas d'infraction et de permettre à l'autorité académique d'enjoindre aux parents de rescolariser leurs enfants lorsque l'établissement fonctionne malgré un refus administratif ou lorsque c'est un établissement clandestin. d'une innovation majeure, et je veux de nouveau saluer l'initiative de Françoise Gatel sur ce point. La nouvelle rédaction proposée par cet amendement vise à simplifier la procédure et à la rendre plus opérationnelle et sécurisante pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées. J'y suis donc favorable.

Celui-ci, constatant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation, pourra, dans l'intérêt de l'ordre public, s'opposer à ce qu'il ouvre ou dirige tout établissement scolaire privé. Le constat s'exercera précisément parce que le bulletin numéro 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l'est déjà sur le fondement de l'article 776 du code de procédure pénale. En revanche, la loi ne peut pas exiger d'une personne qu'elle remette son bulletin numéro 2 ; en effet, l'article 776 du code de procédure pénale ne permet pas à une personne d'obtenir ce document. Un citoyen ne peut obtenir que son bulletin n° 3, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 777-2 et 774 du code de procédure pénale.

à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou dirige un établissement est dans l'illégalité en créant une troisième sanction pénale pour interdire à l'intéressé de diriger ou d'enseigner dans un établissement scolaire, et donc d'ouvrir un tel établissement. le sous-amendement n° 45 rectifié que nous examinerons à l'article 3, prend en compte la nouvelle architecture choisie par la rapporteur et qui a été reprise par l'amendement n° . S'inspirant de la rédaction de l'article 227-17-1 du code pénal, il introduit cette nouvelle sanction aux articles L. 441-4 et L. 914-5 nouveaux du code de l'éducation en cas d'ouverture ou de direction d'un établissement dans des conditions illégales.

C'est là toute la stratégie : dénaturer un dispositif afin d'adopter un texte qui finit par être totalement inefficient. Pourquoi ce sous-amendement- j'emploierai une expression un peu triviale -dézingue-t-il votre proposition de loi, madame Gatel ? Toute personne malintentionnée désirant se soustraire aux conditions d'ouverture déposera intentionnellement une demande d'ouverture incomplète, de préférence concernant l'objet de l'enseignement, et tablera sur les délais d'examen des dossiers par l'administration pour s'exonérer des conditions d'ouverture gênantes pour son projet, et ce d'autant plus que le délai outrancièrement minimaliste de quinze jours est, si je puis m'exprimer ainsi, du pain béni pour les futurs contrevenants.

il répond à la volonté des centristes de faire en sorte que, dans notre pays, la loi puisse être appliquée, que le maire de Raismes, dans le Nord, ne se retrouve pas seul dans un désert de responsabilités et qu'on puisse protéger les enfants de France. Monsieur Assouline, si vous avez des choses à dire sur les positions

Il y a suffisamment de risques de voir se multiplier dans notre pays des structures pseudo-éducatives, qui ont d'autres orientations que celles de partager nos valeurs et de former la libre conscience et le haut niveau d'indépendance intellectuelle et morale de nos enfants,

progresser la protection des enfants au travers de cette proposition de loi, se trouver bizarrement mis en accusation de ne pas vouloir cette protection. Nous sommes tous

Madame Gatel, je répète que nous ne doutons pas de votre volonté ferme ni de votre bonne foi pour mieux encadrer l'ouverture des écoles privées hors contrat dans le pays. Dès lors, pourquoi ne plus faire mention du projet pédagogique, des programmes et des horaires dans les pièces à fournir pour toute ouverture d'établissement, quel que soit le niveau ? N'est-ce donc pas d'école qu'il s'agit, d'instruction, de formation des esprits, d'éducation ? Vous ne pouvez pas considérer que le projet pédagogique, les programmes et les horaires sont des informations insignifiantes ou subalternes pour l'ouverture d'un établissement scolaire privé- ou public, d'ailleurs, si la question se posait. Avoir pour seule référence un objet d'enseignement conforme au socle commun de compétences et de connaissances ne permet pas

Oui à la liberté pédagogique, non à la liberté des programmes que revendiquaient nos collègues du groupe Les Républicains dans leur amendement initial ! Vous êtes très exigeant sur les fondamentaux quand il s'agit de l'enseignement public, et c'est normal

voulant retourner dans l'enseignement public, échouer aux tests de compétences et de connaissances, parce qu'ils auront reçu un enseignement lacunaire ou parcellaire, voire orienté. Nous regrettons

ou association, à n'importe quel moment ? La liberté, c'est, bien sûr, une liberté dans un cadre collectif. Par ailleurs, la première liberté à préserver, c'est celle des enfants.

outre les incapacités visées à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, il convient de mentionner explicitement l'interdiction pour toute personne signalée à l'administration pour des antécédents judiciaires d'entretenir tout lien avec un établissement d'enseignement privé. Il s'agit donc d'élargir

Cet amendement est satisfait par l'article L. 911-5 du code de l'éducation, en vertu duquel sont incapables de diriger un établissement scolaire, d'y enseigner ou d'y être employées les personnes ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs, celles qui ont été privées par jugement de tout ou partie de leurs droits civils, civiques et de famille ou qui ont été déchues de l'autorité parentale et celles qui ont été frappées d'interdiction définitive d'enseigner. De plus, l'amendement fait référence à l'article 706-47-4 du code de procédure pénale. Or l'article 3 du décret du 18 mai 2016 prévoit déjà que les personnes exerçant une activité dans une école privée

aux valeurs qui nous sont communes ne seront pas capables de donner les gages attendus, lors tant de la constitution des dossiers de déclaration d'ouverture que des contrôles. En la matière, je parle d'expérience ... Pour réaliser ces contrôles, indispensables, je le répète, et dont le premier doit être opéré dans la première année qui suit l'ouverture de l'école, les inspecteurs qui en sont chargés doivent être formés à déjouer les multiples opérations de dissimulation des dérives que cette proposition de loi vise à juste titre à combattre. Ce n'est pas toujours le cas. la mission des corps d'inspection doit donc être clarifiée et précisée. Là aussi, des progrès doivent être accomplis, ce qui n'enlève rien au professionnalisme de ceux qui mènent ces missions difficiles. Il y faut une volonté politique, que vous avez exprimée il y a quelques instants, des moyens spécifiques et un vrai plan de formation des personnels. Dans chaque département, un travail collaboratif entre les services de l'éducation nationale

de leurs encadrants est assurée ; que les lois de notre pays visant à la protection de l'enfance et de la jeunesse sont respectées ; que l'organisation des enseignements et leur progression permettent d'atteindre les résultats académiques et les objectifs finaux communs à tous. En revanche, le renforcement des contrôles, que j'approuve, ne doit pas déboucher sur la mise en adéquation forcée de pratiques pédagogiques choisies librement par les écoles hors contrat avec les approches de l'éducation nationale et de ses corps d'inspection, telles qu'elles prévalent dans les établissements publics ou privés sous contrat. Il y a là un véritable risque

l'amendement de rédaction de l'article 2 présenté par Mme la rapporteur en commission. En particulier, il instaure un principe de communication annuelle des informations concernant les enseignants à l'administration de l'éducation nationale,

aux amendements n 31 et 33, ainsi qu'au sous-amendement n° 39 rectifié. L'amendement n° 31 de M. Magner est similaire à l'amendement n° 33 de Mme Gatel. Il en diffère toutefois sur deux points. Il tend tout d'abord à préciser que le contrôle des services de l'éducation nationale peut être « inopiné

entre des centaines de contrôles obligatoires, qui s'ajouteront aux contrôles requis en cas de signalement ou de demande de passage sous contrat, je préfère que les recteurs puissent concentrer leurs moyens sur les établissements qu'ils estiment prioritaires.

le code du travail et le code de l'éducation imposent déjà aux établissements de tenir un registre. Il s'agira simplement d'en adresser chaque année un extrait à l'autorité académique. Par ailleurs, prévoir l'obligation, pour les services de l'éducation nationale, de contrôler les établissements privés au cours de leur première année de fonctionnement, c'est donner force de loi à une prescription qui leur est déjà faite. Les auditions menées par la rapporteur, ainsi qu'une étude effectuée auprès des recteurs et reprise dans le rapport de Mme Billon, traduisent les progrès massifs des services de l'éducation nationale sur la question des contrôles.

qui souhaitent étendre l'obligation de contrôle aux troisième et cinquième années d'exercice des établissements. Faisons pleinement confiance aux inspecteurs de l'éducation nationale pour détecter les établissements problématiques lors du contrôle qu'ils effectueront dès la première année. S'ils estiment devoir y retourner dès la première année, voire la deuxième année, ils pourront

Antoine Karam, pour explication de vote. Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, je suis personnellement très attaché au contrôle des établissements privés hors contrat.

un commerce ; faisons au moins en sorte qu'il soit plus facile de la fermer que de fermer un commerce

Je vous remercie

à instaurer l'interdiction, pour toute personne ayant fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'accueil de mineurs, de diriger un établissement d'enseignement privé ou d'y enseigner. Il s'agit de procéder à un alignement sur les dispositions qui régissent les personnels enseignants de

harmoniser les conditions d'exercice pour diriger un établissement scolaire privé ou y enseigner. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 32, lui préférant l'amendement n° 34 rectifié de Mme Gatel, qui est plus complet. En effet, ce dernier tend à limiter les conditions pouvant être requises pour exercer dans l'enseignement privé en faisant référence aux conditions d'emploi des contractuels de l'éducation nationale. Il prévoit une procédure de sanction spécifique en cas de manquement à cette disposition, contrairement à l'amendement n° 32. l'application de son dispositif ne remettra pas en cause les situations acquises, ce qui est conforme au principe de non-rétroactivité de la loi. La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n°

911-5 du code de l'éducation. Ce dernier exclut en effet de tout emploi dans une école ceux qui ont subi une « condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs », qui ont été « privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille » ou qui ont été « déchus de l'autorité parentale

Le constat s'exercera précisément parce que le bulletin numéro 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l'est déjà sur le fondement de l'article 776 du code de procédure pénale.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article pose la condition d'une récidive dans l'année pour que le tribunal correctionnel puisse prononcer la fermeture d'un établissement scolaire d'enseignement général dont le directeur s'oppose à l'inspection.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à relever la peine prévue à l'encontre des directeurs d'établissement privé hors contrat lorsqu'ils n'ont pas mis en conformité

vise à porter les peines encourues en cas de refus de dispenser un enseignement conforme à l'instruction obligatoire à deux ans d'emprisonnement et à 50 000 euros d'amende. Les six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende prévus me semblent

n° 24 rectifié , le texte de Mme Gatel vise déjà à aligner l'ensemble des peines pénales liées à l'exercice d'activités délictueuses au regard du code de l'éducation dans un établissement scolaire. Cet alignement s'effectue déjà à la hausse sur la peine de 15 000 euros d'amende qui préexiste, notamment en cas d'obstruction à l'inspection dans un établissement technique. Comme pour l'amendement n° 23 rectifié, le relèvement du montant de l'amende à 50 000 euros et la création d'une peine de prison

Mme Françoise Laborde. Cet amendement vise à prévoir un délai de six mois pour permettre aux établissements privés hors contrat déjà ouverts de se conformer aux dispositions prévues par la présente Nous pensons notamment aux conditions d'âge et de qualification et à la communication des noms et des titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement.

en donnant six mois aux établissements déjà ouverts pour s'y conformer. La commission a préféré en rester au principe de non-rétroactivité des lois, afin de ne pas mettre en cause des situations acquises, dans un souci de sécurité juridique. L'avis est donc défavorable. Quel est

et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

et à un renforcement des contrôles. Dans cette perspective, le texte aurait dû, selon nous, répondre à plusieurs conditions cumulatives. Il aurait dû prévoir, comme c'était le cas initialement, l'inclusion du projet pédagogique dans le dossier de déclaration.

Nous voulions rendre obligatoires les contrôles non seulement la première année d'exercice, mais également la troisième et la cinquième années, une demande de contractualisation avec l'État échéance. Nous ne cautionnons pas du tout le délai de quinze jours au terme duquel le dossier de déclaration est réputé complet et la déclaration validée. Pour nous, ce point est totalement inacceptable. À nos yeux, la première liberté à préserver, c'est bien celle de l'enfant : la liberté d'accéder à un haut niveau d'éducation, respectueux des principes républicains Or, nous le constatons, les conditions requises ne sont pas réunies ce soir. Le texte issu du compromis passé entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement, s'il permet quelques avancées en termes d'harmonisation des procédures

La proposition de loi instaure un juste équilibre entre une liberté fondamentale, celle de l'enseignement, et le nécessaire encadrement du régime d'ouverture des établissements.

un net progrès en termes de protection des enfants et de moyens donnés aux autorités pour faire respecter l'obligation d'éducation, dans un cadre de liberté de choix pour les parents. Chacun a affirmé ses principes.

proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Union Centriste. Il va être procédé au